L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2019, Nous poursuivons l'examen, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, des différentes missions.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en 2019, les crédits de la mission « Travail et emploi » s'élèveront à 13,4 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 12,4 milliards d'euros en crédits de paiement.

À cet égard, la contribution de la mission « Travail et emploi » et de ses opérateurs à cet effort est, il est vrai, significative. Les effectifs de la mission diminueront ainsi de 233 équivalents temps plein, permettant une économie, hors pensions, de plus de 5 millions d'euros. Le montant des subventions pour charges de service public versées aux opérateurs sera également en baisse, de plus de 86 millions d'euros, et leurs plafonds d'emplois connaîtront une diminution sensible de 458 équivalents temps plein travaillé. L'essentiel de l'effort demandé aux opérateurs sera porté par Pôle emploi. S'agissant des crédits, cette diminution sera plus que compensée par une hausse de la contribution de l'assurance chômage. Néanmoins, si le nombre de demandeurs d'emploi devait progresser, ou si les missions confiées à l'opérateur dans le cadre de la future réforme de l'assurance chômage devaient s'accroître, il conviendrait sans doute de réexaminer la pertinence de la poursuite de la baisse des effectifs envisagée par le Gouvernement. La diminution des crédits de la mission « Travail et emploi » ne se fait en outre pas à l'aveugle. Elle poursuit une logique de recentrage des moyens sur les publics les plus éloignés de l'emploi. Moins nombreux, les contrats aidés ont vocation à devenir de véritables outils d'insertion des demandeurs d'emploi. La transformation des contrats d'accompagnement dans l'emploi, les CUI-CAE, en parcours emploi compétences, ou PEC, intervenue en début d'année, participe de cette logique. Certes, les conditions pour y avoir recours sont plus restrictives : elles sont la contrepartie d'exigences plus grandes en matière d'accompagnement et de formation du bénéficiaire.

la baisse des contrats aidés sera en partie compensée par un effort en faveur du secteur de l'insertion par l'activité économique, qui bénéficiera de moyens en hausse de 51 millions d'euros par rapport à 2018, permettant le financement de 5 000 équivalents temps plein supplémentaires. Le présent projet de loi de finances porte également l'ambition de construire une « société de compétences ». Sur la durée du quinquennat, un effort inédit sera consenti dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, plan favorisera la formation et l'accompagnement des jeunes et les demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché du travail. Au total, le PIC sera doté de 15 milliards d'euros, parmi lesquels 13,8 milliards d'euros seront portés par la mission « Travail et emploi

Ces crédits budgétaires seront en outre complétés par un fonds de concours de 1,5 milliard d'euros versé par France compétences. Mes chers collègues, le budget qui nous est présenté est donc un budget responsable, dont les orientations sont claires : mieux accompagner les personnes les plus en difficulté et investir dans l'avenir. Aussi, je vous propose d'adopter les crédits de la mission « Travail et emploi », sous réserve de l'adoption déposé avec ma collègue rapporteur spécial Sophie Taillé-Polian, visant à renforcer les crédits consacrés aux maisons de l'emploi. Très bonne chose ! Je vous propose en outre d'adopter les crédits du compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » sans modification. La parole

cette baisse a été rappelée par mon collègue Emmanuel Capus : 500 millions d'euros en autorisations d'engagement et 3 milliards d'euros en crédits de paiement. Certes, le taux de chômage diminue. Cela signifie-t-il pour autant que la situation de l'emploi s'est améliorée au cours des derniers mois ? Rien n'est moins évident. Le nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois en catégorie A a bien diminué entre le premier trimestre 2015 et le troisième trimestre 2018, cette baisse a été plus que compensée par une progression du nombre de demandeurs d'emploi en catégories B et C, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi ayant exercé une activité réduite. En outre, le chômage des plus de 50 ans a progressé de 3 % sur un an, toutes catégories confondues, et de près de 9 % pour les seules catégories B et C. Dès lors, la logique baissière poursuivie par le Gouvernement se fera au détriment des personnes les plus éloignées de l'emploi, comme en témoigne la diminution drastique de l'enveloppe des contrats aidés.

L'argument selon lequel le taux d'insertion dans l'emploi à la sortie d'un contrat aidé était faible ne tient pas, dans la mesure où les bénéficiaires sont précisément les personnes les plus éloignées du marché du travail.

L'augmentation des moyens consacrés à l'insertion par l'activité économique, présentée comme la contrepartie de la réduction de l'enveloppe des contrats aidés, est positive. Néanmoins, l'insertion par l'activité économique ne doit pas être mise en concurrence avec les contrats aidés

S'agissant du plan d'investissement dans les compétences, présenté comme l'innovation majeure de ce gouvernement en matière de politique de l'emploi, je rappelle qu'une part importante des crédits qui lui seront dévolus en 2019 était déjà inscrite dans le budget de la mission « Travail et emploi ». Cela était notamment le cas des moyens consacrés à la garantie jeunes, ou du plan « 500 000 formations », auquel a succédé le volet « formation » du PIC. S'agissant plus spécifiquement de la garantie jeunes, il me semble que ce dispositif gagnerait à être assoupli afin, d'une part, de toucher un public plus nombreux et, d'autre part, d'en simplifier la gestion pour les missions locales. Outre une diminution drastique des dépenses d'intervention de la mission, le Gouvernement a également fait le choix d'affaiblir les acteurs de la politique du travail et de l'emploi. Les missions locales voient ainsi leur budget global baisser. À cet égard, la baisse des effectifs du ministère du travail et, notamment, de ceux de l'inspection du travail est un très mauvais signal alors que, d'une part, le travail illégal et la fraude au détachement constituent des enjeux de plus en plus prégnants et que, d'autre part, le droit du travail a fait l'objet de modifications substantielles au cours des années passées qui nécessitent contrôles et accompagnement. Face à ce paradoxe, le ministère répond que, en France, le ratio des salariés par rapport aux agents de contrôle est conforme au standard fixé par l'Organisation internationale du travail. Néanmoins, au regard de la diversité des missions assignées à l'inspection du travail française, cette comparaison a peu de sens. Plus généralement, l'affaiblissement des opérateurs du travail et de l'emploi est symptomatique de la politique de l'offre mise en oeuvre par le gouvernement actuel et entre en contradiction avec la nécessité d'accompagner davantage les publics les plus éloignés de l'emploi, dont le nombre augmente et dont la situation

Si la dématérialisation peut permettre de simplifier certaines procédures, elle peut aussi s'avérer dissuasive pour certains demandeurs d'emploi. On observe également à Pôle emploi une baisse

bénéficiaires, le plan de transformation lancé par la direction générale le 16 octobre dernier ne manquera pas, malheureusement, d'affaiblir encore cet opérateur et risque de se traduire par une baisse de la qualité du service rendu

qui nie la situation de millions de Français pour qui trouver un emploi ne se résume pas au fait de traverser la rue ! Aussi, bien que vous invitant à adopter l'amendement que j'ai signé avec Emmanuel Capus sur les moyens consacrés aux maisons de l'emploi, qui nous semblent des outils intéressants et importants dans bon nombre de territoires, je vous propose, à titre personnel, de rejeter les crédits de la mission « Travail et emploi ». Je vous propose en revanche d'adopter sans modification les crédits du compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ». La parole

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues rapporteurs de la commission des finances, mes chers collègues, alors que la baisse du chômage demeure très lente et fragile, la baisse du budget de la politique de l'emploi ne peut qu'interpeller. cette baisse résulte en partie d'un effet de périmètre. Néanmoins, à périmètre constant, elle s'élèverait tout de même à 2 milliards d'euros, soit une Elle résulte largement de l'extinction, décidée antérieurement, de dispositifs dont l'inefficacité a été démontrée. Le Sénat et ses différentes commissions ont d'ailleurs eu l'occasion d'approuver leur disparition. Elle résulte, ensuite, de la poursuite de la politique amorcée l'année dernière en matière de recours aux contrats aidés. Si nous avons pu regretter la brutalité de cette mesure, je soutiens le recentrage de cet outil sur les publics les plus éloignés de l'emploi.

sans étude d'impact, de relancer l'expérimentation des emplois francs, qui avait pourtant échoué de manière éloquente par le passé. La montée en charge de ce nouveau dispositif expérimental est largement en deçà des objectifs annoncés ; on peut donc légitimement douter de son succès. Le renforcement des crédits en faveur de l'insertion par l'activité économique et des entreprises adaptées doit, en revanche, être salué. Les autres orateurs ne manqueront pas de souligner les efforts demandés à Pôle emploi, aux missions locales ou encore à l'AFPA, alors qu'un service public de l'emploi fort apparaît toujours nécessaire. La formation des jeunes et des demandeurs d'emploi est une nécessité. On ne peut donc qu'approuver le plan d'investissement dans les compétences, qui doit connaître en 2019 sa première année pleine de mise en oeuvre. L'ampleur de cet effort doit néanmoins être relativisée. Le PIC est en effet artificiellement gonflé par l'intégration de dispositifs déjà existants, dont certains étaient d'ailleurs financés par d'autres lignes budgétaires l'année dernière. En outre, le fonds de concours qui doit être apporté par France compétences correspond en fait à une partie des fonds qui étaient déjà collectés par les organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA. Ce n'est qu'en raison d'une réforme de la tuyauterie financière que ces fonds apparaissent cette année dans le budget de l'État. Ce n'est qu'au prix de ces importants biais de présentation que le Gouvernement peut parler d'un effort sans précédent. Enfin, un certain nombre de décrets nécessaires à la mise en oeuvre de la réforme de l'alternance prévue par la loi du 5 septembre 2018 ne sont toujours pas parus. Cela est regrettable pour la sincérité des débats budgétaires, surtout pour les acteurs, qui se trouvent dans une situation de forte incertitude. Malgré ces observations, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Travail et emploi », des articles rattachés, ainsi que du compte d'affectation spéciale « Financement national

Mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera donc en faveur de ce texte, car il contient des avancées réelles, notamment sur les compétences.

préoccupe. La question de l'efficacité du service public de l'emploi reste posée dans notre pays. Nous le savons bien, reprise économique ne rime pas avec embellie de la situation de l'emploi dans tout le pays,

au moins cette année. Les nouvelles modalités de collecte et d'affectation de la contribution des entreprises au financement de la formation professionnelle permettront, certes, d'afficher un fonds abondé à hauteur de 1,5 milliard d'euros en provenance de la future agence France compétences, mais,

Mes chers collègues, il est difficile pour l'ancien vice-président du département du Nord en charge de l'insertion et du RSA que je suis de ne pas digresser un peu pour partager avec vous une analyse plus proche du terrain.

Nous sommes passés en quelques semaines d'un mal du pouvoir d'achat à une rage du pouvoir d'achat. Cette situation appelle aujourd'hui un traitement de fond de la question de l'emploi, du pouvoir d'achat et de la place de la valeur travail dans notre société.

Je suis un peu sorti de mon texte, mais, voyez-vous, nous sommes aussi ici pour sortir des sentiers battus et affirmer nos valeurs ! Je termine, mes chers collègues, en vous indiquant que nous suivrons l'avis du rapporteur de la commission des affaires sociales : nous voterons en faveur de l'adoption des crédits de la mission « Travail et emploi et emploi » et en faveur de l'article 84 réformant les modalités de versement de l'aide aux entreprises au titre du dispositif d'activité partielle, ainsi que de l'article 84 que nos collègues députés ont ajouté au projet initial, portant le financement de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Nous voterons, enfin, en faveur du compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ». Nous sommes heureux de constater un frissonnement

Monsieur le président, madame la ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le développement de l'activité et de l'emploi est au coeur des préoccupations du Gouvernement et de la majorité. Depuis un an, les résultats sont encourageants : baisse de 1,2 % du nombre de chômeurs inscrits en catégorie A et augmentation du taux d'activité, qui s'établit à 72 %. La diminution des crédits de la mission « Travail et emploi », de l'ordre de 496,6 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 2,9 milliards d'euros en crédits de paiement, s'inscrit dans ce contexte d'amélioration globale de la situation de l'emploi et de maîtrise indispensable de la dépense publique.

elle est avant tout liée à la situation actuelle du marché du travail : le nombre de chômeurs diminue, les dépenses aussi. Elle est, par ailleurs, le fruit de la réduction, ou du transfert, de certains dispositifs d'aide à l'embauche

cette mission : elle se subdivise en quatre programmes et un compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

En d'autres termes, l'État participera au fonctionnement de Pôle emploi à hauteur de 1,6 milliard d'euros et au financement du régime de solidarité d'indemnisation du chômage, à travers l'allocation L'action n° 02 consacre son crédit de 2,1 milliards d'euros à l'amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi pour celles et ceux qui en demeurent très éloignés, grâce à une mobilisation territoriale renforcée au travers du fond d'inclusion dans l'emploi ou des outils d'insertion par l'activité économique. L'objectif de l'État est de recentrer ce type de contrats sur les personnes les plus éloignées du marché du travail et non sur les employeurs. Quant aux associations, la transformation du crédit d'impôt sur

la garantie jeunes, les écoles de la deuxième chance, les établissements pour l'insertion dans l'emploi, l'expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » et, enfin, l'aide aux entreprises adaptées qui accueillent des personnes en situation de handicap. Le programme 103 vise à accompagner les mutations économiques et le développement de l'emploi et porte un plan massif de développement des compétences. Sur la durée du quinquennat, 14,6 milliards d'euros seront mobilisés pour accroître les qualifications et donc l'emploi durable,

la simplification de l'accès à la formation grâce à une plateforme numérique qui rend chaque salarié acteur de son parcours professionnel. Le programme 103 finance également le dispositif des emplois francs, expérimenté jusqu'en 2020, 2020, avec 237 millions d'euros en autorisations d'engagement et près de 71 millions d'euros en crédits de paiement, permettant de couvrir le coût de plus de 25 000 contrats. À propos de ce programme, encore, il faut mettre l'accent sur la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et sur le déploiement du plan d'investissement dans les compétences. mobilisera 14 milliards d'euros entre 2018 et 2022 afin d'accompagner la généralisation effective de la garantie jeunes ainsi que le financement des parcours prévus dans le cadre de son volet formation. Le formation. Le programme 111, relatif à l'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail des salariés du secteur concurrentiel, voit, lui aussi, ses crédits réévalués à la hausse afin de financer la formation des conseillers prud'hommes et des défenseurs syndicaux et de renforcer les actions en matière de santé et de sécurité au travail. Son budget prévisionnel pour 2019 s'élève à 88 millions d'euros en crédits de paiement, contre 86,52 millions d'euros en 2018. En revanche, les autorisations d'engagement sont en forte diminution, en raison du renouvellement, en 2018, des conventions triennales 2018-2020 de l'État pour l'Association de gestion du fonds paritaire national et pour les instituts régionaux du travail du travail social. Le programme 155, enfin, voit ses crédits augmenter de 7 millions d'euros pour atteindre la somme de 689 millions d'euros. Pour rappel, il s'agit d'un programme d'appui et de soutien aux politiques publiques, qui porte sur l'ensemble des 9 500 emplois du ministère. Enfin, les recettes du compte d'affection spéciale consacré au développement et à la modernisation de l'apprentissage augmentent de 77 millions d'euros. Il est important de rappeler ici que ce compte disparaîtra l'an prochain en raison de l'entrée en application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de la création de France compétences.

Madame la ministre, monsieur le président, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2019 prévoit une nouvelle baisse des crédits de la mission « Travail et emploi

Ce budget prétend poursuivre la dynamique de transformation des politiques de l'emploi engagée dans la précédente loi de finances, en augmentant notamment l'effort de formation des jeunes et en améliorant l'efficacité des dispositifs d'insertion dans l'emploi des publics fragiles,

en France s'explique notamment par un déficit de compétences, comme l'a souligné un rapport de l'OCDE publié l'année dernière. Le constat est identique s'agissant de Pôle emploi.

à la fin du mois de novembre dernier, lors d'une grève d'ampleur. Ils ont déploré l'augmentation de leur charge de travail, qui risque de les contraindre à recentrer leur activité sur les missions de contrôle, au détriment de l'accompagnement des demandeurs, pourtant essentiel pour favoriser le retour à l'emploi. Ces suppressions de postes vont aussi concerner l'inspection du travail. Madame la ministre, en novembre dernier vous avez présenté un index de l'égalité femmes-hommes permettant d'évaluer les entreprises et de les sanctionner si nécessaire. que cette politique soit efficacement mise en oeuvre, vous avez promis une multiplication par quatre des contrôles menés par l'inspection du travail. Or cette promesse ne pourra en aucun cas être tenue avec des effectifs réduits.

Nous renouvelons notre opposition à cette mesure qui a un impact direct sur les collectivités territoriales, notamment dans les territoires ruraux, et sur les associations, avec pour conséquence un affaiblissement du service public

ou l'accent mis sur le soutien aux entreprises adaptées, dans le cadre de la politique d'emploi des travailleurs handicapés. Ce coup de pouce ne suffit cependant pas à faire oublier l'accumulation de dispositions négatives adoptées par le Gouvernement, qui ont porté atteinte au pouvoir d'achat et aux conditions d'existence des personnes en situation de handicap.

à moindre coût et nous nous opposons à la pratique qui consiste à prendre d'une main pour donner de l'autre, tout en continuant à restreindre globalement les crédits. Alors même que le taux de chômage reste à 9 %, il est inacceptable que le service public de l'emploi soit affaibli afin de réduire les dépenses budgétaires

vous décidez, comme si rien ne se passait, de maintenir vos politiques visant à faire des cadeaux aux plus riches et à imposer l'austérité aux autres ! Oui, il nous faut ramener la paix et la sérénité dans notre pays.

Monsieur le président, madame la ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la mission « Travail et emploi » apparaît comme l'une des grandes sacrifiées du projet de loi de finances pour 2019. Par rapport au budget de l'année précédente, la baisse des crédits consacrés à l'action de l'État en faveur du travail et de l'emploi est drastique : perdant 500 millions d'euros en autorisations d'engagement et 3 milliards d'euros en crédits de paiement, ces pôles de dépenses respectifs s'élèvent péniblement à 13,4 milliards et 12,4 milliards d'euros pour l'année 2019. Malheureusement, ce tournant budgétaire ne résulte pas d'une embellie majeure sur le marché de l'emploi en France. En effet, si l'indicateur de l'INSEE pointe une baisse de 0,5 point du taux de chômage au deuxième trimestre de l'année 2018, ce dernier semble s'être stabilisé à 9,1 % de la population active au troisième trimestre, soit plus de 2 730 000 chômeurs, toujours à la recherche d'un travail dans notre pays. pays. De plus, cet indicateur masque une triste réalité : la précarisation de l'emploi et un éloignement toujours plus important des chômeurs les plus fragiles. En effet, si l'on observe une baisse de 1 % du nombre de chômeurs de catégorie A, A, celle-ci est malheureusement compensée par une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi des catégories B et C, qui exercent une activité réduite. Maîtrise des dépenses publiques oblige, la contribution exigée de la mission « Travail et emploi », et donc, à travers elle, de ses opérateurs, est considérable. Pôle emploi sera la structure la plus touchée, puisqu'elle supporte l'essentiel de la diminution du montant des subventions, avec un effort chiffré à près de 84,7 millions d'euros la ministre, que l'augmentation de la contribution versée par l'UNEDIC et la baisse des effectifs devraient compenser l'impact pour Pôle emploi de ces mesures, mais aucune garantie n'est avancée contre le risque probable d'une dégradation des conditions de travail des agents et donc du service rendu aux demandeurs d'emploi comme aux employeurs. Concernant les emplois aidés, les prévisions budgétaires annoncent une diminution du nombre d'entrées en contrat de 200 000 en 2018 à 100 000 en 2019. Ce dispositif n'a, certes, pas fait la preuve de sa capacité à favoriser à chaque fois un retour à l'emploi,

Dans le même temps, la mission « Travail et emploi » permet de conforter le lancement du grand plan d'investissement dans les compétences, en faveur de la formation et de l'accompagnement de deux millions de jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, afin de les armer pour satisfaire aux nouvelles exigences du monde du travail. les missions locales chargées de la mise en oeuvre de la garantie jeunes verront leur dotation diminuer. C'est incompréhensible ! Il faut opérer un véritable changement d'échelle ! Le combat contre le chômage et la précarisation du travail ne peut être mené exclusivement par l'État de nombreuses politiques territoriales sont d'ores et déjà orchestrées dans nos métropoles comme en milieu rural, où les élus locaux agissent sur le terrain en faveur de l'emploi et des compétences. des initiatives qui fonctionnent ! Le PIC ne saurait atteindre les objectifs qui lui sont fixés sans les fers de lance que représentent ces plateformes locales d'animation et d'ingénierie, que sont les plans locaux pour l'insertion et l'emploi- les PLIE -et les maisons de l'emploi,

nombreux rapports d'évaluation en témoignent. Lieux reconnus d'ingénierie territoriale et de construction collective de l'emploi, les 106 maisons de l'emploi réparties sur le territoire français sont portées par plus de 15 000 communes et plus 1 500 000 entreprises.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, selon les derniers chiffres d'Eurostat, sortis la semaine dernière, le taux de chômage dans la zone euro a poursuivi sa baisse en novembre 2018 pour atteindre 8,1 %. Il est encore de 9,1 % en France, sans compter les emplois précaires, notamment les emplois aidés. Malgré la reprise de l'activité et la baisse du chômage dans notre pays, nous sommes donc loin de la moyenne européenne.

une diminution record de 500 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 3 milliards d'euros en crédits de paiement ! Malgré cette forte baisse, ils sont maintenus à un niveau élevé par rapport à la moyenne des dix dernières années. Je salue les efforts de pédagogie déployés par le rapporteur spécial, M. Emmanuel Capus, qui nous a démontré que cette baisse s'accompagnait d'un recentrage des crédits vers les dispositifs qui fonctionnent vraiment. Tout d'abord, je souhaite revenir sur la diminution de l'enveloppe consacrée aux contrats aidés,

Le temps est venu de recentrer les moyens sur les publics les plus éloignés de l'emploi. Nous saluons ainsi la transformation des contrats d'accompagnement dans l'emploi en parcours emploi compétences, intervenue en début d'année. J'en viens à l'autre point important de cette mission : la lutte contre le chômage des jeunes et l'investissement dans les compétences. L'augmentation significative des crédits consacrés au plan d'investissement dans les compétences, le PIC, permettra d'accompagner la généralisation effective de la garantie jeunes, notamment dans son volet formation. Le chômage des jeunes atteint 20 % dans notre pays, ce n'est pas nouveau, mais c'est inacceptable. Ce sont les générations futures que nous sacrifions L'accent mis sur la formation des jeunes dans ce projet de loi de finances est donc une bonne orientation. Enfin, j'insiste sur la nécessaire territorialisation des politiques de l'emploi. Pour lutter contre le chômage, il faut bien connaître les situations locales ainsi que les bassins d'emploi et déployer une action de proximité. Nous nous interrogeons donc, comme nos collègues, sur la diminution quasi constante

Nous soutiendrons donc l'amendement des rapporteurs spéciaux Emmanuel Capus et Sophie Taillé-Polian destiné à appuyer ces structures. Merci ! Notre groupe est convaincu qu'un tournant des politiques de l'emploi est nécessaire pour faire face aux mutations du monde du travail ; vous l'avez entamé, un regard positif sur votre politique, qui favorise la montée en compétences de l'ensemble des travailleurs tout au long de leur carrière, l'adaptation rapide aux transformations technologiques et la revalorisation de l'apprentissage, que l'on évoque depuis longtemps et qui est essentielle. Nous voterons ces crédits en l'état, car ils annoncent un redéploiement pertinent des efforts financiers de l'État vers les dispositifs les plus efficaces

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, investir dans les politiques publiques de l'emploi est capital pour permettre à chacun de nos concitoyens, notamment aux plus fragiles d'entre eux, de s'émanciper par le travail. les crédits consacrés à la politique de l'emploi dans le projet de loi de finances pour 2019 vont, malheureusement, à rebours de cette ambition. Pour la deuxième année consécutive, nous assistons à une baisse du budget de 3 milliards d'euros, alors que les derniers chiffres montrent un ralentissement des créations d'emploi et l'échec du Gouvernement à résorber le chômage en 2018. Certes, un effort est tout de même consenti en faveur des structures de l'insertion par l'activité économique, ou encore, s'agissant de l'insertion professionnelle des jeunes, des établissements Ces écoles offrent aux décrocheurs une réelle opportunité de se relancer : 60 % des jeunes passés dans ces structures en sortent avec une qualification ou un emploi.

D'autres dispositifs subissent malheureusement une contraction inexpliquée de leurs moyens. D'abord, le sort réservé aux missions locales suscite l'inquiétude dans nos territoires. En effet, alors que les missions locales sont en première ligne pour la mobilisation de la garantie jeunes,

Une telle décision aurait immanquablement mis ces structures en difficulté, alors même qu'elles interviennent dans des domaines qui ne sont pas toujours couverts par les services publics de l'emploi. Pour une fois, l'Assemblée nationale n'est pas restée sourde à ce sujet : elle a adopté un premier amendement prévoyant une dotation de 5 millions d'euros, complété par un autre amendement, portant sur 10 millions d'euros, proposé par les rapporteurs de la commission des finances du Sénat. Le nouveau montant permettra un soutien effectif de ces structures et évitera le saupoudrage des crédits. L'importante contraction des crédits de la mission est également l'une des conséquences les plus visibles du coup de frein brutal porté à la politique des contrats aidés à l'automne 2017. Moins d'un an après sa mise en place, la nouvelle formule de contrats aidés, les parcours emploi compétences, dits PEC, présente un bilan plus que mitigé. Si l'on observe une sous-consommation des PEC depuis le début de cette année, c'est en partie dû à l'excessive complexité du dispositif. Le coût s'est également avéré dissuasif pour les associations et les petites collectivités territoriales, puisque le taux de prise en charge par l'État a été ramené de 73 % en 2017 à 50 % en 2018. Ajoutons que la diminution du nombre de contrats aidés est intervenue dans un contexte financier déjà fragilisé pour les associations et les collectivités territoriales, en raison de la suppression de la réserve parlementaire et de la baisse des dotations de l'État. Je rappelle que nous ne sommes pas hostiles à l'évolution des contrats aidés vers davantage d'accompagnement et de formation des bénéficiaires. Ce que nous dénonçons, c'est la brutalité avec laquelle cette réforme a été menée. Et quelle réponse pour les petites communes qui n'ont pas les moyens d'embaucher autrement ? Aucune solution alternative ne leur a été apportée au budget de Pôle emploi, il en baisse de 85 millions d'euros, après une baisse de 50 millions d'euros en 2018. Là encore, j'ai du mal à comprendre ce choix : ce n'est pas en réduisant les moyens humains et financiers de Pôle emploi et en augmentant dans le même temps les charges des conseillers- 70 dossiers supplémentaires pour chacun avec le plan pauvreté -que la situation des demandeurs d'emploi s'améliorera. C'est une aberration, car nombre de personnes ont plutôt besoin d'être prises par la main. permettez-moi d'aborder la question du handicap. S'il faut saluer l'effort de 15 millions d'euros portant à 400 millions d'euros au total les financements en faveur de l'emploi des personnes handicapées, beaucoup reste à faire pour améliorer leur situation. la prise en charge de la prestation de compensation du handicap, la PCH, reste insuffisante pour ceux qui travaillent et doivent financer les équipements nécessaires pour s'adapter à leur emploi, comme un véhicule adapté ou un fauteuil. On constate aussi de nombreux retards dans le paiement des aides, et l'expérimentation en cours visant à faire prendre en charge la PCH par les fonds départementaux de compensation du handicap s'avère complexe, en raison des finances exsangues des départements. Madame la ministre, nous souhaitons le meilleur pour la France. Chaque fois qu'une bonne mesure en faveur de l'emploi est proposée, nous la votons sans hésitation, comme nous l'avons fait avec les ordonnances Travail. faut conclure. Je m'y emploie, monsieur le président. Malgré les nombreux points négatifs de ce budget et faute de pouvoir majorer les crédits, nous voterons tout de même en faveur de cette mission, pour les quelques avancées qu'elle comporte. Mais quelle déception pour les Français éloignés de l'emploi ! La parole est

Monsieur le président, madame la ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la lutte contre l'exclusion et le chômage exige des politiques d'insertion professionnelle fortes et ambitieuses. D'autant plus quand les chiffres du chômage ne sont pas bons, malheureusement. Or, d'après les dernières statistiques de la DARES, toutes catégories confondues, la France compte plus de 5 600 000 demandeurs d'emploi. Un chiffre tristement en hausse, sur trois mois comme sur un an. pour la deuxième année consécutive, le budget de la mission « Travail et emploi » est marqué par une forte contraction des crédits de paiement, qui s'établissent à 12,4 milliards d'euros, soit 3 milliards d'euros de moins qu'en 2018, à périmètre comparable. En pratique, on assiste à un affaiblissement des différents opérateurs du travail et de l'emploi, particulièrement symptomatique de la politique mise en oeuvre par le Gouvernement, en totale contradiction avec la nécessité d'accompagner davantage les publics les plus fragilisés et éloignés de l'emploi. L'opérateur Pôle emploi est particulièrement touché, avec une baisse de sa subvention pour charges de service public à hauteur de près de 85 millions d'euros, qui fait suite à la baisse de 50 millions d'euros intervenue cette année. Les effectifs de Pôle emploi vont être durement touchés. D'ores et déjà, une baisse de 800 équivalents temps plein est annoncée pour l'an prochain, sans tenir compte du redéploiement de certains conseillers vers l'activité de contrôle. En 2018, près de 500 postes et 1 000 contrats aidés ont déjà été supprimés. À Pôle emploi comme ailleurs, on justifie ces coupes par des gains de productivité- encore évoqués il y a quelques instants -, qui reposeraient notamment sur le tout-numérique. Or si la dématérialisation peut simplifier les procédures, elle peut aussi s'avérer dissuasive pour certains publics. Rien ne remplace l'écoute et l'accompagnement d'un conseiller ! Derrière tout cela, je vois surtout une dégradation du service public de l'emploi et des conditions de travail des agents, aux portefeuilles de suivi et d'accompagnement toujours plus fournis. Les missions locales, elles aussi, vont être encore fragilisées, par la diminution de plus de 8 millions d'euros des crédits consacrés aux conventions d'objectifs, alors que certaines ont déjà été mises en difficulté par la baisse des subventions des collectivités territoriales, aux budgets toujours plus contraints. Cela correspond à la suppression de 250 emplois de conseiller. Cette baisse de moyens est un paradoxe, au moment où le Gouvernement va confier aux missions locales de nouvelles responsabilités dans la lutte contre la pauvreté des jeunes, notamment avec l'obligation de formation. Quant aux expérimentations des fusions des missions locales dans Pôle emploi, nous y sommes opposés. Elles vont conduire à remettre en cause la spécificité de l'accompagnement global et personnalisé des jeunes, ainsi que l'ancrage territorial des missions locales et l'engagement politique et financier fort des élus représentant leur collectivité Nous considérons que les missions locales doivent conserver leur expertise et continuer à assurer leur rôle de service public territorialisé de l'insertion des jeunes, notamment dans le cadre de la montée en puissance du dispositif garantie jeunes. Concernant les contrats aidés, nous avions dénoncé, l'an passé, la baisse drastique de leur nombre. Force est de constater que les nouveaux parcours emploi compétences

le taux de prise en charge par l'État est trop faible, l'obligation de formation n'est pas financée et vous avez perdu la confiance de nombre d'employeurs, qui redoutent un nouveau revirement du Gouvernement. C'est tout de même un comble que la sous-consommation des contrats aidés en 2018 vous permette de justifier des crédits et un nombre d'entrées en contrat encore en baisse pour 2019 vous disiez vouloir privilégier le qualitatif par rapport au quantitatif. Au bout du compte, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Les emplois aidés manquent notamment dans les services scolaires et périscolaires, dans l'aide aux personnes dépendantes, dans les EHPAD et, tout aussi cruellement, dans le milieu associatif. Les conséquences en sont dramatiques dans nos territoires.

Que dire de la disparition dans ce projet de loi de finances de la contribution de l'État au budget de fonctionnement des maisons de l'emploi ? Elle mettra inexorablement en difficulté ces structures. Je crains que seules quelques collectivités territoriales ne soient en mesure de conserver leur maison de l'emploi, et qu'on ne laisse de côté les demandeurs d'emploi des zones déjà défavorisées. Si l'amendement adopté par l'Assemblée nationale visant à consacrer une enveloppe de 5 millions d'euros aux maisons de l'emploi va dans le bon sens, ce montant reste insuffisant. C'est pourquoi notre groupe défendra un amendement visant à porter ces crédits à 10 millions d'euros. Madame la ministre, la diminution des effectifs de votre propre ministère, notamment de ceux de l'inspection du travail, est un très mauvais signal, à une époque marquée par des modifications substantielles du droit du travail et alors que la lutte contre le travail illégal devrait vous préoccuper. Pour toutes ces raisons, et bien que les mesures en faveur de l'insertion professionnelle

L'analyse de leurs effets nécessitera quelque temps, mais je crains un manque d'anticipation de ces effets sur les entreprises adaptées et les établissements d'aide par le travail. La sous-traitance et les prestations ne pourront pas, à l'avenir, être autant mobilisées qu'aujourd'hui par les employeurs pour s'acquitter partiellement de leur OETH. Il paraît paradoxal d'augmenter si fortement la création de postes, notamment au sein des entreprises adaptées, quand, en même temps, il y a un véritable risque de diminution de leurs carnets de commandes, par l'application des nouvelles règles de calcul de l'OETH. De plus, malgré les nombreuses annonces gouvernementales exhortant à décloisonner et à fluidifier les parcours des personnes handicapées, on peine encore à penser le travail de ces dernières en dehors d'une étanche tripartition entre milieu protégé, milieu adapté et milieu ordinaire. Or il est impossible de modifier l'équilibre de l'un de ces milieux sans bouleverser celui des autres et, par ricochet, affecter les travailleurs qui y sont employés. Pour que les mesures que vous proposez, madame la ministre, soient véritablement efficaces pour l'emploi des travailleurs handicapés, il conviendrait de compléter la réglementation pour permettre à ceux-ci de passer plus facilement du milieu protégé au milieu ordinaire, d'une place dans un établissement médico-social à un emploi au sein d'une entreprise. concerne l'insertion par l'activité économique, l'augmentation des crédits de la mission permettra également la création de 5 000 équivalents temps plein supplémentaires. On ne peut que saluer cet effort, mais il ne compensera que partiellement la diminution importante des emplois aidés. importante des emplois aidés. En ma qualité de membre du conseil d'administration du fonds de l'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, je voudrais présenter les résultats intermédiaires de cette opération. À la suite de l'adoption de la loi du 29 février 2016, dix territoires, dont celui de Mauléon, dans les Deux-Sèvres, ont été sélectionnés afin de tester ce dispositif innovant. Un premier bilan intermédiaire laisse apparaître des résultats très encourageants. Ainsi, au 30 juin dernier, après dix-huit mois d'expérimentation, sur l'ensemble des dix territoires, près de 1 000 personnes ont été recrutées sur un emploi pérenne. Les entreprises à but d'emploi ont créé des emplois supplémentaires non concurrents et utiles. Le 13 septembre dernier, à l'occasion de la présentation du plan contre la pauvreté, le Président de la République a annoncé sa volonté d'étendre cette expérimentation à quarante nouveaux territoires. J'aimerais, madame la ministre, que vous nous indiquiez les conditions dans lesquelles cette expérimentation sera étendue. Aujourd'hui, on dénombre un certain nombre d'outils pour l'insertion par l'activité économique, destinés notamment à aider les personnes éloignées de l'emploi de l'emploi : les parcours emploi compétences, les ateliers et chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion, les entreprises à but d'emploi, les entreprises adaptées, etc. Peut-être serait-il utile de donner une meilleure lisibilité et une certaine cohérence à l'ensemble de ces dispositifs, qui restent efficaces et nécessaires. nécessaires. Est-ce là la future mission du service public de l'insertion annoncé dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté ? Madame la ministre, le Gouvernement se veut actif en matière de lutte contre le chômage, mais, aujourd'hui, les effets durables de la politique menée

Alors que l'ensemble des territoires étaient couverts, ces fermetures de site priveront onze départements des services de l'AFPA, ce qui nuira une fois de plus- c'est une habitude avec ce gouvernement -aux plus fragiles de nos concitoyens et aux territoires ruraux. On assiste à un affaiblissement d'un opérateur historique de la formation professionnelle, alors même, madame la ministre, que vous prétendez faire de la formation professionnelle votre priorité. Le groupe socialiste et républicain défendra un amendement tendant à abonder les crédits budgétaires en faveur de l'AFPA. Car l'affaiblissement de cet organisme profiterait au secteur privé, qui ne pourrait pas forcément fournir un service de qualité. Malheureusement, il y a là une nouvelle illustration du double langage du Gouvernement : vous annoncez des objectifs qui paraissent, parfois, louables, mais vous mettez concrètement en place des politiques qui ne correspondent pas aux effets d'annonce. D'où le sentiment, chez une large majorité de nos concitoyens, d'être trompés.

Cette aide unique est ciblée sur les entreprises de moins de 250 salariés et sur les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat. Cette simplification nécessaire pour les entreprises concernées était attendue, mais, sachant qu'il reviendra au Gouvernement de fixer le montant de l'aide unique par décret, la vigilance s'impose concerne les crédits budgétaires consacrés à l'insertion par l'activité économique, après une forte mobilisation des acteurs du secteur l'année dernière, une augmentation de 5 000 équivalents temps plein est

Enfin, je veux, à mon tour, mettre l'accent sur la catastrophe que représente pour mon département du Pas-de-Calais la suppression des emplois aidés. Avec ce vaste plan de licenciements, vous avez, madame la ministre, augmenté le chômage, donc la souffrance sociale. Par idéologie, vous avez provoqué des catastrophes sociales sur nos territoires, en particulier sur les plus fragiles. Les emplois aidés manquent dans les EHPAD pour nos aînés, manquent aux associations qui se voient affaiblies. Notre tissu social est fragilisé, les solidarités sont entamées, et le sentiment d'abandon de nos concitoyens augmente cruellement : on en voit pour partie la traduction dans les mouvements de protestation actuels. je veux me faire le porte-parole des souffrances de nos concitoyens, qui perçoivent de plus en plus les injustices de votre politique. Le Gouvernement n'écoute pas, il est sourd, campé dans ses certitudes, face à la colère du peuple, alors que votre système ne marche pas, puisque le chômage ne diminue pas, voire progresse. Votre politique de l'emploi n'ayant pas de résultats, il est logique que les sénateurs socialistes et républicains s'y opposent résolument, en particulier en votant contre les crédits de la mission « Travail et emploi » pour 2019 ! La parole

résolus. Bien sûr, les orientations du Gouvernement ont en grande partie été prises précédemment, à l'occasion des ordonnances Travail et de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Force est de reconnaître que de nombreux points allaient dans le bon sens. Adapter les compétences aux mutations que nous connaissons, économiques, sociales ou technologiques, était nécessaire. Seulement voilà : contrairement à ce que l'exécutif laisse entendre, le chômage n'a pas baissé. Selon l'INSEE, le taux de chômage au troisième trimestre de 2018 était stable, à 9,1 % de la population active en France entière.

Pourtant, les budgets alloués à la formation et au travail sont importants, même si une baisse de 2,9 milliards d'euros est prévue pour l'année prochaine, pour une meilleure maîtrise de la dépense publique. Depuis des années, nous critiquons les budgets affectés aux formations et aux différents outils existants, car nous n'avons aucun retour sur les résultats obtenus en matière de lutte contre la précarité. Lutter contre le chômage des jeunes et des personnes les plus éloignées du travail reste une priorité. je suis favorable à la reconduction des crédits destinés à la garantie jeunes, à la reconduction des crédits alloués aux écoles de la deuxième chance et aux établissements pour l'insertion dans l'emploi, aux crédits consacrés au plan d'investissement dans les compétences et à l'insertion par l'activité économique. En revanche, je regrette la diminution de 4 % des moyens alloués aux missions locales, qui oeuvrent concrètement et font un véritable travail de terrain pour répondre aux défis de l'emploi de manière circonstanciée, sur leur territoire. Ces structures associatives accueillent plus de 1,4 million de jeunes chaque année, avec des résultats positifs, puisque près d'un jeune sur deux s'est vu proposer un emploi ou une formation. formation. Elles risquent aujourd'hui l'asphyxie financière et d'être phagocytées par Pôle emploi. Pôle emploi doit aussi connaître une baisse de ses effectifs, compensée par une meilleure productivité. Permettez-moi d'en douter ... Si Pôle emploi reste la structure reconnue par tous, ce n'est plus l'axe privilégié par les employeurs en recherche de salariés. Avec la sur-administration imposée, Pôle emploi ne peut exercer pleinement son activité principale et doit à tout prix se réformer pour confier la gestion des jeunes aux missions locales et aux organismes de réinsertion celle des personnes éloignées de l'emploi. Je pense que l'administration imposée à Pôle emploi n'est pas toujours nécessaire et qu'elle peut être revue pour permettre aux fonctionnaires d'exercer pleinement leur activité de recherche d'emplois. Actuellement, bon nombre de demandeurs d'emploi sont envoyés vers des formations sans débouchés sans débouchés ou qui ne sont pas suivies, afin que les bénéficiaires ne perdent pas leurs avantages. Pendant ce temps, des emplois ne sont toujours pas pourvus ! La politique en matière d'emplois est aujourd'hui beaucoup trop laxiste, malgré des budgets importants. Il est urgent que des comptes soient rendus pour estimer les outils mis en place, leur coût et leur efficacité. Je suis convaincu que nous pouvons mieux faire, avec moins de moyens. Enfin, je regrette aussi la diminution des contrats aidés, qui ont permis à des jeunes en situation de précarité d'intégrer des collectivités territoriales pour être formés et, à terme, employés. Certes, cela représente un coût pour l'État, mais une personne au chômage coûte aussi cher, même si ce ne sont pas les mêmes budgets. le ministre, il est indispensable que la politique du travail et de l'emploi soit revue pour que les demandeurs d'emploi n'hésitent plus à reprendre le chemin du travail et que les emplois soient dorénavant pourvus

Tout d'abord, au-delà de nos convergences et, sur certains points, de nos divergences, je tiens à souligner que vos interventions, en séance comme en commission, témoignent d'une volonté que nous partageons pleinement : permettre à l'ensemble de nos concitoyens, quels que soient leurs origines, leur lieu de résidence et leur parcours, d'accéder à un emploi durable et de qualité. Tel est le sens du cap fixé par le Président de la République et de la politique mise en oeuvre par notre gouvernement : l'émancipation par le travail et la formation. 2019, nous poursuivrons la transformation profonde des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle que j'ai engagée dès mon arrivée, en parallèle des ordonnances pour le renforcement du dialogue social.

Les chantiers ont été nombreux, à commencer par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette loi réforme les règles de gouvernance et de financement des politiques de formation professionnelle et d'apprentissage, avec un remettre l'individu au centre du jeu, en position de décideur, d'acteur de son propre parcours et permettre un développement massif de l'apprentissage, une meilleure efficacité de la formation professionnelle continue, une meilleure inclusion dans l'emploi des personnes en situation de handicap et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. D'autre part, elle élargit la couverture de l'assurance chômage pour faciliter les transitions professionnelles, lutter contre la précarité et asseoir le retour à l'emploi durable. Ces objectifs sont au coeur du document de cadrage remis aux partenaires sociaux en septembre dernier. réponse à vos questions, je confirme que l'ensemble des décrets d'application seront publiés au plus tard début janvier ; plusieurs l'ont déjà été. Par ailleurs, l'ensemble des acteurs opérationnels ont déjà été informés du contenu de ces décrets pour que les délais de procédure ne les empêchent pas d'anticiper sur leur mise en oeuvre.

Le premier objectif, qui est le principal, est évidemment de faire en sorte d'accompagner et de former les personnes peu qualifiées, jeunes sans qualification ou demandeurs d'emploi de longue durée, dans une logique d'acquisition de compétences très attendues sur le marché du travail.

aidés précédent en contrats aidés parcours emploi compétences. La dimension territoriale du pilotage de ces outils d'insertion a été renforcée avec la création du fonds d'inclusion dans l'emploi, qui permet une fongibilité et une adaptation locale aux moyens en fonction des besoins observés. Le quatrième chantier engagé a trait au renforcement sans précédent du modèle inclusif des entreprises adaptées pour les personnes en situation de handicap. C'est le sens de l'accord pluriannuel « Cap vers l'entreprise inclusive 2018-2022 » que j'ai signé avec le secteur

Toujours en 2018, un plan de transformation de l'AFPA a été annoncé il y a quelques semaines, mais nous y reviendrons plus tard dans le débat. Je tiens à souligner que l'ensemble de ces actions ont été menées dans le respect du plafond des crédits qui m'ont été alloués. souligné, le budget de la mission « Travail et emploi » est de 12,4 milliards d'euros. À périmètre constant, il y a bien une baisse de crédits de 2 milliards d'euros par rapport à 2018, mais cette baisse est liée, en quasi-totalité, à deux facteurs. Le premier, c'est l'extinction, décidée par le précédent gouvernement, des mesures dont j'ai pris acte à mon arrivée, à savoir la suppression de l'aide ponctuelle à l'embauche des TPE et PME.

Ce budget poursuit les efforts engagés en 2018 avec deux objectifs très clairement affirmés, qui en sont la colonne vertébrale. Il s'agit d'abord de l'investissement dans les compétences du développement de tous les dispositifs d'inclusion dans l'emploi pour les plus vulnérables, en cherchant à chaque fois le plus efficace au service de nos concitoyens. Il est primordial que les personnes les plus vulnérables soient replacées au coeur des politiques d'inclusion. Cela fait partie de l'objectif visé par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, présentée par le Président de la République le 13 septembre dernier. C'est dans cet esprit de transformation et en multipliant les déplacements sur le terrain dans le cadre de la semaine de l'apprentissage, de celle de la lutte contre la pauvreté, ou de mes déplacements hebdomadaires, que j'ai construit le budget de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'exercice 2019. Tout d'abord, je tiens à souligner que nous poursuivrons la montée en puissance du plan d'investissement compétences avec un doublement des crédits alloués. Ce nouvel engagement de 3 milliards d'euros

Ces crédits seront mobilisés selon quatre orientations. Le premier objectif, qui correspond à près de la moitié du plan d'investissement compétences, est la mise en oeuvre des parcours de formation dans le cadre des pactes régionaux pluriannuels d'investissement dans les compétences, qui sont en cours de négociation entre l'État et les régions

est de faire un effort particulier pour certains publics. Je pense notamment aux 60 millions d'euros par an qui seront consacrés à la formation des bénéficiaires de l'insertion par l'activité économique. Ce volet formation manquait souvent

Le plan d'investissement compétences permettra aussi de renforcer les capacités d'accueil dans les écoles de la deuxième chance et l'EPIDE. Le quatrième objectif est de promouvoir les expérimentations fondées sur des approches innovantes portant soit sur des secteurs cibles, soit sur des publics cibles. J'en citerai quelques-unes les 10 000 formations numériques, les 10 000 formations aux emplois verts, mais aussi le plan massif de mobilisation pour le retour à l'emploi dans les QPV, les quartiers prioritaires de la ville,

particulièrement dans les quartiers prioritaires de la ville où l'on constate que les jeunes ont très peu accès à cette voie d'excellence et de réussite. En ce qui concerne les « territoires zéro chômeur », l'évaluation aura lieu. Nous augmentons les moyens

si la deuxième étape de l'expérimentation, plus large, le confirme. S'agissant des personnes en situation de handicap, je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà expliqué en commission.

Le budget de l'emploi pour 2019, au-delà du plan d'investissement compétences, prévoit un engagement important en direction des publics les plus vulnérables.

Comme indiqué précédemment, l'année 2019 sera aussi l'année du plein déploiement de la réforme des entreprises adaptées. Un budget de 400 millions d'euros, en augmentation par rapport à 2018, sera consacré à cette ambition en 2019.

Ces efforts seront complétés par 100 000 nouveaux parcours emploi compétences. Je disais qu'ils correspondent aujourd'hui à la dynamique actuelle. Nous constatons déjà un meilleur ciblage sur les personnes en difficulté et un meilleur taux d'accès à la qualification. 30 000 contrats aidés seront dédiés à l'accompagnement des élèves en situation de handicap à l'école et transférés au budget du ministère de l'éducation nationale, soit 124 millions d'euros de crédits à cet effet.

qui est dynamique, assise sur la masse salariale, augmentera d'environ 100 millions d'euros pour atteindre 3,5 milliards d'euros. Les moyens de Pôle emploi seront donc bien en hausse en 2019.

dans les zones rurales et au bas des tours dans les quartiers prioritaires de la ville. J'ai d'ailleurs créé un conseil de l'inclusion dans l'emploi, présidé par Thibaut Guilluy, pour suivre de façon plus dynamique La réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage se traduit dès le budget sur deux autres aspects : la simplification du paysage des aides à l'apprentissage, et donc une aide unique pour les entreprises dès le 1janvier 2019 pour l'apprentissage, et la création du nouvel opérateur France compétences. En termes de coût du travail, une simplification du paysage des exonérations, avec la bascule de certains allégements spécifiques vers le droit commun, qui s'appliquera dès le 1janvier 2019, le droit commun étant plus favorable que les allégements spécifiques précédents.

Tout cela suppose une meilleure coordination des acteurs au service de l'emploi. Nous y travaillons. Je précise que nous n'envisageons pas une fusion mais une coopération très renforcée, comme nous l'avons fait entre Cap emploi et Pôle emploi cette année.

S'agissant des effectifs du ministère, la baisse sera de 233 emplois, soit un taux d'effort- 2,5 % -stable par rapport à 2018, qui n'empêchera pas la mise en oeuvre de nos missions. Car le ministère relève aussi le défi du numérique et la modernisation du système d'information du ministère en appui des politiques de l'emploi contribue à cette efficacité. En conclusion, j'ai souhaité partager avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs, la grande cohérence de ce budget, qui porte deux grandes ambitions : intensifier l'effort d'inclusion pour favoriser l'émancipation par l'emploi et stimuler la création d'emplois et le développement des emplois par l'investissement dans les compétences, la libération de l'apprentissage et un renforcement de l'effort en matière de baisse du coût du travail. Nous allons

Au second semestre de cette année, ce sont 48 sections d'inspection du travail qui y ont été supprimées. À cela s'ajoute un terrain juridique en perpétuelle évolution qui appelle les inspecteurs à une mise à jour quasi permanente.

touchent à la lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement. Madame la ministre, vous venez de lancer une campagne nationale de sensibilisation au risque de chutes de hauteur, qui figure parmi les priorités du troisième Plan santé au travail. Votre collègue Marlène Schiappa, de son côté, souhaite que les inspecteurs du travail se consacrent au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes par les employeurs. Soit

La rationalisation de l'action autour des priorités 2019 consiste à mettre en place une meilleure priorisation, ce que nous avons commencé à faire en 2018. Nous avons quatre grandes priorités : la lutte contre le travail illégal, la lutte contre la fraude au travail détaché,

rappelle que l'on constate depuis plusieurs années une baisse du nombre d'interventions par inspecteur du travail. Nous voulons retrouver un rythme qui permette une présence moyenne de deux jours par semaine en intervention pour les inspecteurs du travail.

les fraudes au détachement. Ce qui est efficace, et nous le faisons de plus en plus, c'est les interventions conjointes de l'inspection du travail, de la police et la gendarmerie, de l'URSSAF, des services fiscaux, et des douanes.

on arrive à faire beaucoup mieux. C'est là ce que nous voulons faire.

social à l'AFPA. Je l'ai dit précédemment, ce sont onze départements qui se trouveront sans site de service public de formation professionnelle pour adultes. D'ailleurs, les salariés de l'AFPA manifesteront jeudi. Nombre d'élus locaux et de parlementaires de notre groupe s'inquiètent de la fin de ce maillage territorial et de l'avenir des salariés licenciés. Il s'agit d'un service public de proximité en moins dans un contexte où emploi et territoires sont des enjeux majeurs, permet tout de même un taux de retour à l'emploi de 70 %. Dans les Hauts-de-France, ce ne sont pas moins de trois sites qui sont concernés par une fermeture : Berck-sur-mer, Boulogne-sur-mer et Beauvais. De plus, ce sont des centres bien implantés et reconnus, tel que celui d'Agen-Foulayronnes, qui forme près de 400 stagiaires chaque année, dont 60 % de chômeurs, et qui constitue un centre référent dans le domaine du froid. Les salariés de l'AFPA ne comprennent pas que l'on ferme des formations qui affichent complet, telles que la formation de technicien de maintenance climatique et énergies renouvelables ou certaines formations dans des secteurs sous tension comme la restauration. Je rappellerai que nous ne sommes pas restés inactifs pour sauver l'AFPA, puisque nous avons opéré un plan de refondation stratégique au cours des années 2014 à 2017, qui a permis une progression sur les marchés avec les entreprises, et a abouti à la transformation de l'agence en EPIC. Cet amendement est avant tout un amendement d'appel, en particulier sur l'avenir des personnels licenciés. Quel

avec les caractéristiques économiques du territoire. Les témoignages sont nombreux pour souligner à quel point l'AFPA est une chance, notamment pour les personnes éloignées du marché du travail, qui reprennent ainsi pied et construisent leur parcours de réinsertion. L'annonce de la suppression du centre de l'AFPA de Nevers a donc été un réel choc. Elle a suscité beaucoup d'incompréhension dans la Nièvre, mais aussi dans le Cher et dans l'Allier. Pour le seul centre de Nevers, ce sont dix-sept contrats à durée indéterminée qui sont menacés de suppression et plusieurs milliers d'heures de formation qui risquent d'être perdues. La fermeture de ce

de redonner du souffle aux personnes concernées. Madame la ministre, nous avons déjà eu ce débat et je vous demande, à l'image de ce que réclament nos concitoyens, de nous écouter, d'entendre ces craintes légitimes et d'agir dans l'intérêt de tous les territoires, de tous les habitants et de tous les chômeurs. Contraindre les gens à parcourir plusieurs kilomètres pour trouver un autre centre de formation, ce n'est pas un bon signal donné à nos concitoyens ! Fermer un centre de formation qui fonctionne et dans lequel de gros investissements ont été réalisés sur les plateaux techniques, ce n'est pas juste ! Prendre la décision de supprimer dix-sept contrats à durée indéterminée, alors que

de cette antenne. Les Nivernais n'en étant pas responsables, ils n'ont pas à en subir les conséquences ! La parole

concernés par l'expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée », lancée sous le quinquennat de François Hollande. Il s'agit d'une excellente mesure pour réinsérer professionnellement des personnes durablement éloignées de l'emploi, tout en répondant à des besoins des populations non couverts par le marché, par la construction concomitante d'une offre de service territoriale. Au 30 juin dernier, après deux ans d'expérimentation

et l'objectif totalement rempli. À Colombelles, dans mon département, le Calvados, l'expérience menée est également très positive et concluante. Malheureusement, à ce stade, le doublement du nombre de chômeurs concernés par ce dispositif s'apparente

Le président du fonds d'expérimentation, Louis Gallois, estime, lui-même, que l'expérimentation est suffisamment concluante pour pouvoir être développée sur de nouveaux territoires. Avec cet amendement, il s'agit de prendre le Gouvernement au mot, en doublant dès maintenant le nombre de personnes remises au travail le programme « Territoires zéro chômeur de longue durée », et, ainsi, de répondre aux territoires en attente de développer des entreprises à but d'emploi- ou EBE -dans le cadre de l'extension de cette expérimentation.

Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail, de 14,07 millions d'euros,

des aspects -, sur le plan humain, des hommes et des femmes relèvent la tête, participent à la vie de la cité, dans des associations, à l'occasion d'événements, etc. Ils ont retrouvé leur dignité

Plusieurs collègues se sont également exprimés pour défendre le rôle de ces maisons de l'emploi et de la formation dans notre maillage territorial. L'État, en abandonnant ces structures, laisse les collectivités se débrouiller avec cette mission, si essentielle, que représente l'insertion professionnelle des jeunes. Cet abandon des maisons de l'emploi et de la formation est d'autant plus incompréhensible que le Président de la République s'est engagé à multiplier par cinq l'accueil des jeunes dans le cadre du plan Pauvreté présenté voilà deux mois.

Depuis un an, madame le ministre, je vous demande audience en tant que présidente des maisons de l'emploi, pour vous parler de cet outil, né des territoires, de la volonté d'élus qui oeuvrent pour l'emploi et l'insertion. Depuis 2005, date de leur création par Jean-Louis Borloo, les maisons de l'emploi ont adapté leurs missions aux évolutions des territoires et des besoins sociétaux, en lien avec chaque ministre successif du travail et de l'emploi.

Elles sont aussi le support de clauses d'insertion, ce dispositif selon lequel 72 % des personnes les plus éloignées de l'emploi restent en CDI après dix-huit mois de contrat. C'est le dispositif le plus évalué, et toujours positivement

le mépris pour un outil auquel ils sont attachés. Le Sénat se mobilise, sur toutes les travées, pour vous demander des crédits supplémentaires. Merci de l'entendre, madame la ministre.

dans ce budget pour 2019. Les maisons de l'emploi permettent de faire le lien entre les différents partenaires publics et privés, d'élaborer une stratégie au niveau local et de développer l'emploi. Le retrait des financements de l'État est particulièrement dommageable pour les collectivités qui sont dans une situation financière difficile, car elles ne pourront plus financer ces maisons de l'emploi. Cette mesure aggravera donc les inégalités territoriales. C'est la double peine pour les habitants de ces territoires, privés d'emploi et de structures d'accès à l'emploi ! Vous le savez, mes chers collègues, notre pays connaît un taux de chômage élevé, puisqu'il s'établit à 9 %- 11,7 dans ma région, les Hauts-de-France, dont le taux de pauvreté atteint 18 %, plus de 20 % dans mon département du Pas-de-Calais. Pourtant, ce projet de loi de finances organise un recul global du service public de l'emploi, et un certain nombre d'opérateurs essentiels

Nous nous opposons à cette politique par laquelle l'État se désengage des initiatives en faveur de l'emploi. Il est nécessaire de maintenir un service public de l'emploi de proximité accessible pour tous, sur tout le territoire. Pour ces raisons, nous proposons de rétablir les financements des maisons de l'emploi. La parole

à l'activité indispensable des maisons de l'emploi sur nos territoires. Dans mon département, notamment, je tiens à souligner le dynamisme dont fait preuve la maison de l'emploi et de la formation de Mulhouse sud-Alsace pour répondre aux besoins des entreprises et des actifs et contribuer à la lutte contre le chômage. Qu'il s'agisse de l'anticipation des mutations économiques, du développement de l'emploi local, de l'orientation ou de la mise en oeuvre du plan local pour l'insertion et l'emploi, ou PLIE, les équipes sont toujours à pied d'oeuvre. Ainsi, sur mon territoire, les maisons de l'emploi ont largement contribué au succès des clauses sociales d'insertion dans les marchés publics. Elles ont également oeuvré au développement de l'emploi et de l'apprentissage transfrontaliers. je mentionnerai une implication dans le travail de fond sur la promotion des mobilités professionnelles pour tous les actifs, dans la droite ligne de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, que nous avons adoptée cette année. Ce réseau mérite donc tout notre soutien. La parole

Entre les fermetures de sites de l'AFPA, la fusion des missions locales avec Pôle emploi et le désengagement de l'État dans les maisons de l'emploi, c'est tout le service public de la formation et de l'emploi dans nos territoires qui est rogné ! Or nous avons besoin de structures de proximité. Cette réduction du périmètre et de l'efficacité des structures territoriales publiques de l'emploi inquiète fortement les élus locaux impliqués dans cette politique publique de toute première importance pour nos concitoyens. Je pense en particulier, sur mon territoire, à la maison de l'emploi et de la formation de l'agglomération caennaise, la MEFAC. Je pense à sa présidente, pour qui le changement d'échelle entraîné par le plan d'investissement compétences, le PIC ne pourra se faire sans l'implication et la mobilisation des plateformes locales d'animation et d'ingénierie que sont les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les maisons de l'emploi. Dans le même esprit, le rapport de la mission d'information du Sénat relative aux maisons de l'emploi a conclu à un bilan gain-efficacité négatif,

Ainsi le plan Pauvreté vise-t-il un quintuplement du nombre de bénéficiaires de la garantie jeunes. Or le présent projet de loi de finances ne fixe comme objectif que 100 000 nouveaux jeunes entrants pour 2019, ce qui est notoirement insuffisant et en contradiction avec l'affichage du Gouvernement. Il convient donc de renforcer la capacité d'accompagnement des jeunes en difficulté par les missions locales, parce que la garantie jeunes ne se résume pas à une simple allocation, mais intègre un volet accompagnement. C'est d'ailleurs ce qui a fait le succès et l'efficacité de ce dispositif. S'il est bien prévu une augmentation de 40,4 millions d'euros des crédits du financement de l'allocation de la garantie jeunes, d'abord, celle-ci est liée à la capacité des missions locales de répondre à des appels à projets dans le cadre du Fonds social européen, et, ensuite, rien n'est prévu en matière d'accompagnement de ces jeunes par les missions locales. Pis, les crédits dédiés à l'accompagnement de tous les jeunes, hors garantie jeunes donc, soit tout de même 86,4 % des jeunes, diminuent fortement, ce qui remet en cause la capacité d'information, d'orientation pour une prise en charge la plus adaptée et l'accompagnement de l'ensemble des jeunes en difficulté d'insertion professionnelle. Ce à quoi il convient d'ajouter une perte de 250 équivalents temps plein. Le Gouvernement se prive ainsi d'une réelle capacité à lutter contre les 20 % de jeunes non diplômés qui vivent sous le seuil de pauvreté et dont le taux de chômage atteint 56 %. Nous vous demandons, madame la ministre, de la cohérence dans votre politique et de sortir des effets d'annonce en maintenant le financement des missions locales à son niveau

émet un avis défavorable sur cet amendement qui vise à augmenter de 8,3 millions d'euros les crédits pour les conventions pluriannuelles d'objectifs conclues avec les missions locales.

madame la ministre. et sa participation est dynamique. Ce financement est triple : un financement structurel ; un financement au titre des missions d'accompagnement exercées par la garantie jeunes ; un financement pour le développement du parrainage. Si l'on considère ces trois enveloppes, le financement global des missions locales par l'État

que d'avoir trois enveloppes différentes faisant l'objet de trois conventions et de trois négociations, nous souhaitons une globalisation des crédits versés aux missions locales pour tirer les conséquences de l'intégration durable de la garantie jeunes dans leur offre de service et leur permettre d'avoir plus de souplesse de gestion. C'est évidemment un aspect dont nous souhaitons discuter aussi avec les collectivités territoriales,

Elle masque la réalité des moyens dévolus aux missions locales, qui, au titre des conventions pluriannuelles d'objectifs conclues avec l'État, vont perdre 8,2 millions d'euros, alors qu'elles ont la charge de la montée en puissance de la garantie jeunes. L'annonce du plan Pauvreté, la volonté du Gouvernement de faire bénéficier de ce dispositif 100 000 jeunes supplémentaires n'est donc qu'un écran de fumée. Madame la rapporteur l'a justement dit dans son intervention : la garantie jeunes est un système très complexe à mettre en oeuvre, tant dans ses obligations de résultat, excessives, que dans ses modalités d'évaluation, inadaptées.

Au final, elles ne perçoivent en moyenne que 85 % des financements : ce ne sont donc pas 1 600 euros qu'elles touchent par jeune, mais 85 % de 1 600 euros. Il faut simplifier cette bureaucratie excessive et non pas supprimer les crédits. S'agit-il là d'affaiblir ces opérateurs de l'emploi, pourtant reconnus, pourtant spécialisés, pourtant de proximité ? S'agit-il de les affaiblir encore et encore, afin de montrer qu'ils n'ont pas la capacité de réaliser cette prise en charge des jeunes ? Que se passera-t-il ?, ?, le Gouvernement justifiera la rationalisation des dispositifs, annoncera ou, en tout cas, favorisera leur fusion avec Pôle emploi. On connaît la méthode Terrible erreur ! Les élus sur l'ensemble de nos territoires y sont fermement opposés. La preuve : quand M. le Premier ministre a fait cette annonce brutale, sans concertation préalable, en juillet dernier, c'est à une véritable levée de boucliers qu'il s'est confronté. C'est devenu alors une expérimentation, annoncée dans le cadre du plan de transformation Action publique 2022. Il faut se méfier de cette expérimentation : les missions locales ne font pas le même métier que Pôle emploi. Il faudrait que les élus maintiennent leur contribution financière

À ce propos, si la concertation est établie avec les professionnels pour s'assurer que l'application réponde bien aux besoins des acteurs privés du marché de la formation, une telle concertation est-elle envisagée en direction des usagers de cette future application ?

Vous nous répondrez sans doute qu'un financement complémentaire est prévu le PIC, mais nous n'avons aucune garantie sur ce point ni aucune information sur son montant. D'où notre amendement. Quel

et de la modernisation de l'apprentissage », figurant à l'état D. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets aux voix ces crédits. Nous avons

Merci